L'exonération de ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers ne doit toutefois pas se faire par une augmentation du ticket modérateur sur les transports programmés.

Alors que 3 millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens ne disposent pas d'une complémentaire santé, cette augmentation est une double peine. Monsieur le ministre, j'en profite pour attirer votre attention sur notre débat concernant le reste à charge. Vous vous êtes réjoui, dans une précédente intervention, du fait que le reste à charge restait de 6 % à 7 % depuis plusieurs années. Mais je veux insister sur un élément qui me paraît extrêmement important : la prise en charge ne se fait pas sur les dépassements d'honoraires. Et j'attire votre attention, notamment, sur les restes à charge

En effet, le Gouvernement compte équilibrer financièrement le coût de l'article 21, qui prévoit la prise en charge intégrale des transports urgents préhospitaliers, par une augmentation du ticket modérateur sur les transports pour soins programmés, renvoyant la prise en charge de cette augmentation

définitive, de l'accès à une couverture complémentaire. Des mesures ont été adoptées l'année dernière pour favoriser l'accès à la complémentaire santé solidaire, qui permet de couvrir sans coût, ou du moins à moindre coût, les personnes à faibles revenus. Une grande campagne de communication a été récemment lancée par le Gouvernement et par l'assurance maladie pour faire bénéficier les patients les plus démunis de cette complémentaire santé solidaire, qui prendra en charge cette

démagogiques, au fantasme de la solution miracle qui émergerait soudain après des décennies d'errance et de turpitudes concernant les déserts médicaux. Voilà quelques décennies ont été prises par par le Parlement de mauvaises décisions, pourtant issues de cerveaux intelligents, des décisions dont les Françaises et les Français paient encore aujourd'hui les conséquences : je veux parler de décisions de régulation de l'offre de soins, donc de régulation du nombre de médecins, ce fameux auquel, je m'en souviens, les professionnels de santé étaient opposés- ils étaient même descendus dans la rue Comment pouvait-on imaginer qu'en limitant le nombre de médecins on allait faire disparaître les besoins de santé dans une population que l'on savait déjà vieillissante ? Et pourtant, ceux qui prirent cette décision étaient sûrs d'eux

Car utiliser la coercition et contraindre ou interdire l'installation de médecins libéraux serait au mieux contre-productif et, quoi qu'il en soit, dégraderait certainement encore davantage la situation des déserts médicaux. Des solutions existent pour lutter contre ces déserts médicaux ; elles sont dans ce PLFSS et dans l'action que je mène et vais continuer de mener. Je vais les exposer brièvement. Auparavant, sans prétendre être Nostradamus, je peux vous prédire ce qui va se passer si vous décidez de prendre la voie de la coercition mes jeunes collègues ne choisiront plus la médecine générale ; de peur d'être obligés d'aller travailler où ils ne veulent pas, ils choisiront une autre spécialité. Et, quand bien même ils choisiraient cette spécialité de médecine générale ou où la coercition s'adresserait à toutes les spécialités, ils choisiront un exercice salarié, en ville, sans contraintes, et s'occuperont de moins de patients ou se limiteront, comme cela se fait de plus en plus, à des centres de soins immédiats non programmés, négation de la médecine du médecin traitant. Comment ferait-on peser sur les jeunes générations seules les erreurs passées ? La pénurie de médecins touchant de nombreux pays, nos jeunes médecins, dont la formation est reconnue au niveau international, quitte à ne pas s'installer où ils le souhaitent, seront tentés d'exercer à l'étranger. La tentation est forte, en effet, et les filières sont en train de se recréer, avec le Canada, l'Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse, ainsi que, très récemment, les Émirats arabes unis, qui proposent aux jeunes médecins généralistes un salaire de 25 000 euros par mois.

Il n'y a pas de solution miracle. Pourtant, mesdames, messieurs les sénateurs, des solutions existent. Il faut avoir le courage de faire les bons choix, des choix d'avenir, des choix susceptibles de refonder notre système de santé dans son ensemble, des choix permettant de voir plus loin que la prochaine échéance.

c'est simplifier les démarches bureaucratiques, chronophages et souvent inutiles. Promouvoir l'installation dans certains territoires, c'est simplifier cette installation par un guichet unique et faire découvrir ces territoires aux jeunes médecins dans le cadre de la quatrième année, professionnalisante, de médecine générale, mais aussi, dès le début de leurs études, dans le cadre de stages ambulatoires. ne nous dise pas que nous manquons de maîtres de stage : nous en aurons 14 000 l'année prochaine ! Faciliter l'exercice médical avancé en favorisant les consultations dans les territoires sous-dotés par des médecins de zones moins démunies,

territoriales, financières ou sociales, c'est refonder notre système sur la réponse aux besoins de santé de la population et non plus sur une logique mortifère d'offre de soins. C'est construire à partir des territoires, avec les Français et les élus, en faisant confiance aux professionnels. C'est tout sauf une politique coercitive, verticale, en définitive inefficace et même dangereuse. C'est au contraire l'esprit de cette refondation que nous devons réussir ensemble dans le cadre du Conseil national de la refondation. Oui, le Gouvernement veut faire confiance aux Français, aux professionnels de santé et aux élus. C'est avec optimisme, mais sans naïveté, que je poursuis cette quête. C'est là tout l'esprit de l'article 22 que nous vous proposons : ce dispositif permet, en cas d'échec, de revenir sur la méthode dans le cadre de la discussion conventionnelle avec les médecins, selon la logique de droits et de devoirs partagée par tous. céder à la facilité, comme quand en 2003 on a accepté de revenir sur l'obligation de garde, que tant de territoires regrettent aujourd'hui. Très bien ! Ce serait une provocation envers les médecins libéraux et la garantie d'une dégradation rapide et durable du dialogue social, d'une dégradation de l'offre de soins et d'une dégradation des soins eux-mêmes. J'ai consulté l'ensemble des organisations syndicales de médecins : elles y sont toutes défavorables. Je sais que l'impatience est grande et que, partant, la tentation est forte d'aller vers la simplicité, voire le simplisme. Mais la santé des Françaises et des Français doit-elle reposer sur une intuition ou sur une politique cohérente, construite avec des arguments irréfutables et bâtie sur une coconstruction avec toutes les parties prenantes ? La balle est dans votre camp, mesdames, messieurs les sénateurs ; s'il vous plaît, ne marquez pas contre votre propre équipe, l'équipe France !

Mme Raymonde Poncet Monge. Certaines personnes, en activité professionnelle et ayant besoin de soins, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d'activité professionnelle délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive. C'est le cas par exemple de certaines personnes dialysées et souhaitant maintenir leur activité professionnelle : il peut arriver qu'elles se rendent dans un centre pratiquant la dialyse après les heures de travail, centre qui peut se trouver

de favoriser le maintien en emploi. Par ailleurs, certaines personnes en situation de handicap se voient dans l'obligation de se rendre dans un centre de soins plus éloigné de leur domicile, mais plus adapté à leur handicap. Or ces personnes se voient refuser la prise en charge au motif qu'il existe un centre situé plus proche que des personnes à mobilité réduite ne disposant pas d'un moyen de locomotion renoncent à des soins non pris en compte dans le cadre d'une ALD, tels que des rendez-vous chez le dentiste, du fait d'une absence de prise en charge des transports dans ce cadre. Certains patients se voient également refuser des prises en charge par des centres de soins ou des professionnels de santé et sont dans l'obligation de s'éloigner de leur domicile. Cet amendement vise donc à permettre la prise en charge des frais de transport dans toutes les situations nécessaires, afin de lever les difficultés d'accès aux soins. Quel est l'avis

De nombreuses situations peuvent déjà conduire à la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport nécessaires pour recevoir des soins ou des examens appropriés à son état de santé : il existe d'ores et déjà onze motifs de prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport sanitaire. Des travaux sont en cours pour améliorer la prise en charge du transport de personnes en situation d'obésité et la Cnam engage des réflexions pour mieux adapter la prise en charge des transports des personnes en situation de handicap. Compte tenu de ces éléments, j'émets un avis défavorable sur cet amendement. La parole est à Mme

par « capitation ». Cette tarification spécifique repose sur un forfait versé aux établissements en fonction du nombre de patients qu'ils accueillent et de leur typologie : âge, sexe, Que le patient vienne consulter une fois, dix fois ou vingt fois dans l'année, le forfait restera identique. L'objectif : inciter les médecins à mettre l'accent sur la prévention et limiter les prescriptions de soins abusives. Mais la tarification à la capitation porte un défaut intrinsèque : le tri des patients. Ce nouveau mode de rémunération pourrait permettre de fidéliser des patients « rentables » dès leur arrivée dans un centre de soins primaires, tandis que les patients les plus « coûteux » seraient réorientés vers l'hôpital. Pour rappel, Ramsay est un mastodonte qui engloutit des cliniques privées : en douze ans, Ramsay Santé est devenu le numéro un de l'hospitalisation privée par le nombre d'établissements. Il représente près de 21 % des parts de marché de l'hospitalisation privée en France, pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 milliards d'euros en juin 2021, soit le double de celui de 2011 ! Ramsay Health Care est par ailleurs coté en Bourse à Sydney, sa valeur étant estimée à 12,2 milliards d'euros. La tentative de racheter les centres de santé détenus par par la Croix-Rouge a échoué, mais l'inquiétude demeure quant à l'arrivée et au développement de cet acteur à but lucratif dans le secteur des soins primaires. Cet exemple est emblématique : quand le service public est mis à mal, faute de financement, quand il est abandonné, cela laisse la place au privé et à toutes les dérives afférentes- je pense aux cabinets de conseil qui pénètrent le secteur de la santé, ou encore à la « licorne » Doctolib. Parce que, Parce que, plus de trois ans après son adoption, on voit bien que cet article 51 entraîne des dérives, nous demandons son abrogation. Quel est l'avis de

sur l'application de cet article. Quelque 1 073 projets ont été déposés depuis 2018. Sur les 494 dossiers recevables, 67 sont en cours d'instruction

Le financement à l'épisode de soins a du sens ; une expérimentation a été menée par exemple sur un tel financement pour des prises en charge chirurgicales dans onze régions. Nous le savons, le mode de financement de notre système de soins doit évoluer ; cela est valable en ville comme à l'hôpital. Or, pour faire évoluer un système, il faut savoir expérimenter

il est hors de question qu'elle soit pérennisée et systématisée. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Mme la rapporteure, mais plus d'un million de patients bénéficient de ces expérimentations, qui sont indispensables si l'on veut faire avancer notre système de santé.

Cet article nous a semblé assez emblématique du manque d'ambition de ce texte. Si le Gouvernement indique qu'il souhaite « rénover la vie conventionnelle », l'article 22 ne modifie en réalité qu'à la marge les règles entourant la négociation des conventions professionnelles entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Ces conventions, qui fixent les conditions de rémunération et d'exercice, constituent pourtant un enjeu essentiel. Une mesure mérite toutefois d'être signalée : vous le savez, l'article 22 ajoute à la liste des thèmes entrant dans le périmètre des négociations conventionnelles de l'ensemble des professions de santé le conventionnement dit « conditionnel Il faut préciser néanmoins que ces dispositions ne contraignent pas les partenaires conventionnels à adopter une mesure en ce sens et, surtout, n'autorisent pas non plus le Gouvernement à le faire de manière unilatérale. s'inscrit dans un contexte particulier : des négociations entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins doivent s'ouvrir et permettre la conclusion au premier trimestre 2023 d'une nouvelle convention médicale, qui définira les conditions d'exercice et de rémunération des médecins pour les cinq prochaines années. Parce qu'il lui a paru souhaitable de permettre aux partenaires conventionnels de s'emparer de ce sujet, la commission vous proposera de conserver les dispositions permettant d'inscrire le conventionnement conditionnel à l'ordre du jour des négociations. que des mesures structurantes ne sauraient résulter que du dialogue avec les organisations représentatives et avec les ordres professionnels ; elle croit en l'esprit de responsabilité de chacun, au service de l'accès aux soins de tous les Français. Ce n'est pas en prenant des mesures coercitives quand la démographie médicale est basse que nous réglerons les problèmes d'accès aux soins. La parole sur l'article. L'article 22 met à jour les dispositions légales qui encadrent les conventions passées entre l'assurance maladie et les professions de santé. Il fait ainsi apparaître pour la première fois, parmi les conditions à remplir par les professionnels pour être conventionnés, leur présence ou non dans les zones sous-dotées. En résumé, on pourrait ouvrir la porte à un conventionnement sélectif, alors même que les jeunes- cela a été dit -ne sont pour rien dans la situation actuelle.

On a applaudi les médecins lorsqu'ils se sont mobilisés pendant la crise ; on les applaudit chaque fois qu'ils répondent présent, comme ces dernières semaines avec l'épidémie de bronchiolite. Les applaudir, c'est bien ; les écouter, c'est mieux. Ils ont des propositions à faire, mais n'approuvent pas ces mesures qui consistent à faire peser sur leurs épaules des décennies de politiques de santé qui nous ont conduits dans cette situation. Plus on contraindra, moins le métier sera attractif. Attention aux solutions simplistes quand le problème est complexe ! C'est une politique générale d'attractivité des territoires et des métiers qui nous permettra, dans l'attente de l'augmentation des effectifs tant attendue après la suppression du, de résorber le phénomène de la désertification médicale.

Cet article prévoit de compléter la liste des thèmes qui peuvent être abordés dans toutes les conventions professionnelles en y ajoutant en particulier « les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones » sous-dotées, mais également « les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé ». Cette disposition constitue, ni plus ni moins, une mesure de coercition déguisée ; la régulation à l'installation ne réglera en rien les problèmes d'accès aux soins.

inspiré des propositions du groupe de travail transpartisan sur les zones sous-denses vise à flécher l'installation des médecins généralistes et spécialistes vers les zones où l'offre de soins est particulièrement faible

que si et seulement si elles sont accompagnées de mesures structurelles en faveur de la diversification de l'origine sociale et surtout géographique des étudiants en médecine,

peuvent permettre d'assurer le service à la population, bien que sur un temps limité. Ainsi, avec cet amendement, nous proposons un premier pas vers la régulation de l'installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de réduire la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées.

Alors que l'actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu'à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux- mesures que nous soutenons, mais qui montrent aujourd'hui leurs limites -, le candidat Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur d'une régulation de l'installation des médecins indiquant ceci le 17 mars dernier : « Ce vers quoi je souhaite qu'on avance, c'est de stopper les conventionnements dans les zones qu'on considère comme déjà bien dotées. C'est un mécanisme qui est efficace. » La régulation de l'installation des médecins est en effet un système qui a montré son efficacité pour d'autres professionnels de santé en France- infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes -et pour les médecins à l'étranger, notamment en Allemagne. Depuis la réélection du Président de la République, cet engagement semble toutefois avoir disparu. Si le présent article prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé et l'assurance maladie, il n'apporte aucune garantie qu'un tel mécanisme soit instauré, ce qui n'est pas satisfaisant. Aussi, cet amendement vise à prévoir que dans les zones surdotées identifiées par les agences régionales de santé un nouveau médecin ne peut s'installer en étant conventionné que lorsqu'un médecin de la même zone cesse son activité ou s'il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone sous-dotée. Les trois

Face à l'urgence à lutter contre les inégalités d'accès aux soins, une politique de maillage du territoire d'offre de soins de premier recours est indispensable.

matière de santé. Ainsi, les personnes pauvres ont trois fois plus de risques que les autres de renoncer à des soins. Si ces personnes se situent en zone sous-dotées, le risque est plus de huit fois supérieur pour le reste de la population. Cependant, l'accès aux soins ne peut pas se résumer à la médecine de ville ; la crise de l'hôpital joue aussi un rôle déterminant dans la progression des déserts médicaux. Les fermetures des hôpitaux, de maternités et plus généralement de lieux de santé de proximité ont précipité l'extension des déserts médicaux. Cet amendement, présenté par notre groupe depuis près de dix ans, vise donc à instaurer un conventionnement sélectif à l'installation dans les zones à forte densité médicale. Nous proposons un mécanisme qui limite l'installation des médecins au départ d'un médecin de cette même zone. Nous nous félicitons de constater que d'autres groupes politiques déposent désormais au Sénat et à l'Assemblée nationale le même type d'amendement. L'amendement

M. Jean-Luc Fichet. Au-delà de l'année de professionnalisation et dès l'obtention du diplôme, il s'agit de conditionner la signature de la convention prévue par l'article L. 162-5 pour un médecin souhaitant exercer dans une zone surdotée à l'exercice de son activité dans une zone dite « normale » d'au moins douze mois en équivalent temps plein sur une période de trois La période est réduite à six mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans dans une zone sous-dotée. Pendant cette durée totale de trois années, les modes d'exercice pourront, bien entendu, être souples- libéral, salarié, temps partagé hôpital-cabinet -pour permettre le travail d'équipe et le contact régulier avec un ou plusieurs confrères référents, remplaçant d'un médecin, adjoint d'un médecin, signataire avec une agence régionale de santé d'un contrat prévu à l'article L. 1435-4-2, salarié d'un médecin libéral ou d'un centre de santé.

les dispositions prévoyant que les partenaires conventionnels peuvent négocier un conventionnement sélectif, au motif que cette solution ne serait pas la bonne. Les suivants visent, au contraire, à l'imposer aux médecins par la loi, sans attendre l'issue des négociations à venir. Le conventionnement sélectif des médecins, et plus largement la répartition des médecins sur le territoire est un sujet important sur lequel nous nous sommes, mes chers collègues, déjà penchés à de nombreuses reprises. Encore récemment, la proposition de loi du président Retailleau, largement reprise par le Gouvernement dans le PLFSS, a été adoptée par le Sénat afin de rendre obligatoire la réalisation par les étudiants de médecine générale d'une quatrième année de stage en priorité en zones sous-dotées. La commission a toutefois jugé qu'il n'était pas souhaitable, alors que s'ouvrent des négociations essentielles en vue d'une nouvelle convention médicale, d'adopter maintenant de nouvelles mesures coercitives. Nous pensons qu'il ne faut ni éluder le sujet en le supprimant des thèmes pouvant être abordés par l'assurance maladie et les syndicats ni court-circuiter les négociations en imposant, dès maintenant, par la loi, des mesures coercitives qui risqueraient d'être mal comprises des professionnels et de décourager les jeunes médecins à s'installer. L'amélioration de l'accès aux soins figure parmi les priorités de l'assurance maladie dans la négociation qui s'ouvre. Elle est bien plus large que le conventionnement sélectif, qui ne réglera rien à lui tout seul : ni les problématiques de temps médical disponible- j'insiste sur ce point sur ce point -, qui requièrent de réfléchir au partage des responsabilités entre professions de santé comme au développement des assistants médicaux ni celles qui sont relatives à la démographie des médecins. Tout au plus, dans le contexte actuel, contribuera-t-il à répartir la pénurie. Convaincue que les mesures coercitives ne sont jamais aussi efficaces que lorsqu'elles ont été négociées, la commission vous propose de laisser les partenaires conventionnels s'emparer de ce sujet comme, plus largement, des questions d'accès aux soins dans les prochains mois, avant d'envisager de légiférer.

La commission souhaite que ces thèmes soient abordés au cours de l'ensemble des négociations à venir. L'amendement n° 883 vise à conditionner l'installation d'un médecin à une autorisation de l'ARS et, dans les zones surdotées, au départ d'un médecin. Je crains que ce type de mesure ne décourage l'installation alors que nous sommes en situation de pénurie. J'émets donc un avis défavorable. L'amendement n° 13 rectifié tend à subordonner le conventionnement d'un médecin dans une zone surdotée au départ d'un autre médecin ou à l'exercice préalable en zone sous-dotée. Même avis défavorable pour la même raison. 541 rectifié visent à réserver le conventionnement dans les zones surdotées aux médecins de secteur 1, et à subordonner tout nouveau conventionnement au maintien d'une certaine proportion de médecins conventionnés fixée par voie réglementaire et au départ d'un autre médecin.

je ne sais pas ce que cela veut dire, et les ARS non plus d'ailleurs puisqu'elles ne sont pas amenées à définir ce qu'est un territoire surdoté ! Vous évoquez des exemples à l'étranger. En Allemagne, cela aurait réglé le problème : je suis désolé de vous décevoir, c'est faux, cela n'a absolument pas réglé le problème, comme dans tous les pays qui ont voulu mettre en place la coercition, y compris au Canada et au Québec, que l'on cite souvent en exemple. Je vous invite à vous reporter au rapport de la Drees de décembre 2021, qui fait une analyse de toutes les solutions mises en place dans les pays étrangers pour répondre à la désertification médicale. Les solutions proposées sont

jeunes. Ils vont donc, en plus, pouvoir s'enrichir en vendant leur clientèle, alors que les médecins des secteurs les plus difficiles, qui travaillent la nuit, n'auront absolument pas cette possibilité. On crée ainsi une inégalité entre les secteurs et entre les médecins, ce qui pour moi est totalement inacceptable

? Il n'y a pas de solution miracle.

! Des millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Il faut agir, ça n'est pas de la coercition ! Faisons attention aux mots et ne manipulons pas les idées en n'employant pas le bon vocabulaire.

jours est emblématique de l'état de notre société. L'Association des maires ruraux de France a produit moult enquêtes attestant dans quel état se trouvent la plupart de nos communes.

et pas des spécialistes ... Nous devons vraiment faire un effort de réflexion. Monsieur le ministre, je suis d'accord avec mes collègues sur la question de la convention. Il faudra batailler dur

par le marché fait le bien commun. Non, ce n'est pas la réalité ! Et si l'on refuse toute organisation

en ayant expliqué aux médecins que s'ils ont des droits et des envies, ils ont aussi des devoirs, comme nous tous.

Le problème, c'est que l'on manque de médecins : il y a des zones pourvues, des zones insuffisamment pourvues et des zones pas du tout pourvues. Mais il n'y a pas de zones « sur-pourvues

de l'année prochaine ; l'exercice partagé ; les expérimentations d'accès direct de l'article 24 ; l'accroissement du nombre d'assistants médicaux, qui permettent d'augmenter de 10 % la patientèle de chaque médecin, et la simplification de leur mise en place ; le cumul emploi-retraite ; et l'article 25, sur la « libération » des

Mon amendement vise à renforcer le soutien à l'usage des outils numériques en améliorant l'équilibre des différentes aides financières entre professionnels de santé. Le soutien de l'assurance maladie à l'équipement informatique et aux usages des services numériques des médecins libéraux, le forfait structure, est actuellement quatre à huit fois supérieur à celui qui est accordé aux autres professionnels de santé.

et à développer des pratiques coopératives et coordonnées, une telle différence n'encourage malheureusement pas une adhésion égalitaire à l'utilisation de tels outils par les différentes catégories de professionnels de santé. Or les bénéfices du numérique sont incontestables pour les organisations, les professionnels et les citoyens : simplification de l'accès aux soins, développement de nouvelles pratiques à distance, coopération entre les acteurs de la santé et fluidification des parcours de soins. Les travaux engagés dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé ont permis de prendre la mesure de la nécessité d'amélioration sur ce point : des dispositions visant à renforcer les démarches de soutien en faveur des médecins libéraux Afin de soutenir l'usage des outils numériques, il est proposé dans l'amendement d'ajouter à la définition des conventions nationales la prise en compte de l'équilibre des financements visant à investir dans des outils informatiques entre les professionnels de santé. Élargir la définition des dispositions communes aux conventions nationales encouragera l'adhésion des professionnels de santé pour plus d'universalité et de pluridisciplinarité au service des patients. Quel

en temps utile par le Parlement. Pour améliorer le contrôle parlementaire sur les conventions conclues, cet amendement vise à remplacer, dans le code de la sécurité sociale, le délai de six mois nécessaire avant l'entrée en vigueur d'une mesure conventionnelle dépensière par une condition relative à l'adoption d'un projet de loi de financement tenant compte des conséquences des mesures dépensières sur la trajectoire des dépenses d'assurance maladie. Si certaines mesures conventionnelles apparaissent urgentes au Gouvernement, celui-ci sera toujours libre de soumettre au Parlement dans son projet de loi une dérogation ponctuelle à ces dispositions qu'il justifiera dans l'étude d'impact. Quel

dans une loi de financement de la sécurité sociale. L'adoption de l'amendement n° 52 rectifié permettrait au ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une convention

le vote du Parlement et le contenu des conventions. Il s'agit aussi de vous donner les moyens, sous le contrôle du Parlement, de vous assurer que la dimension financière des conventions est prise en compte de manière adéquate par les négociateurs. Ainsi, notre commission se montre cohérente avec ce qu'elle a déjà défendu lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques la semaine dernière. La maîtrise de cette énorme masse de dépenses publiques qu'est l'Ondam ne peut plus s'effectuer, comme par le passé, en faisant payer par l'hôpital année après année le dépassement des dépenses de soins de ville. Il faut donc des outils de régulation. Par cet amendement, nous vous en fournissons Dire cela, ce n'est montrer personne du doigt. C'est simplement une question élémentaire d'équité et de bonne gestion. La situation de l'hôpital ne laisse de toute

la légitimité des syndicats représentatifs. Il convient de rappeler que ces derniers font l'objet d'une enquête de représentativité menée par la direction de la de la sécurité sociale au regard du score obtenu aux élections des unions régionales des professionnels de santé (URPS), de leur présence territoriale, du nombre d'adhérents, de leur autonomie financière et de leur activité en direction de la profession. Il est essentiel que les syndicats professionnels représentatifs demeurent des interlocuteurs incontournables lors des diverses négociations, notamment dans le cadre d'une concertation départementale. La parole est à

Ces derniers font l'objet d'une enquête de représentativité, menée par la direction de la sécurité sociale, au regard du score obtenu aux élections de l'URPS, de leur présence territoriale, du nombre d'adhérents, de leur autonomie financière et de leur activité en direction de la profession.

par les organisations représentatives des professions de santé. Ces dernières estiment que la loi remet en cause leur légitimité à représenter l'ensemble des professionnels en exercice libéral dans les négociations conventionnelles. Par ailleurs, le Gouvernement les a modifiées à l'Assemblée nationale, reconnaissant que la représentation des maisons de santé n'était pas encore suffisamment structurée pour permettre leur participation aux négociations. La mesure apparaît insuffisamment préparée et non concertée avec les organisations représentatives. En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur ces amendements.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements

est ainsi libellé : La parole est à Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à permettre aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une convention dont les conséquences financières remettraient en cause de manière substantielle la trajectoire des dépenses d'assurance maladie votée par le Parlement. La Cour des comptes a relevé, dans le rapport 2022 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, que le coût financier d'une convention ne figurait pas parmi les motifs pouvant justifier une opposition des ministres. Pourtant, les conventions professionnelles constituent un élément structurant des dépenses de soins de ville. Il est nécessaire de mieux anticiper et de mieux suivre leurs conséquences financières. Tel est l'objet de cet amendement.

Les bilans de médication constituent une mission spécifique attribuée aux pharmaciens d'officine, afin de s'assurer de la bonne observance du traitement par le patient et d'éviter la iatrogénie médicamenteuse. Ces interventions pharmaceutiques ne doivent pas être confondues avec des accompagnements se concentrant sur une pathologie spécifique du patient,

par celle d'« entretiens d'accompagnement d'un assuré ». Cette mise à jour est souhaitable pour le suivi des patients atteints d'une pathologie chronique, désormais élargi sous forme d'entretiens d'accompagnement. En revanche, elle ne l'est pour les bilans de médication, qui ne se limitent pas à un entretien, mais s'appuient au contraire sur une suite d'entretiens réguliers avec le patient

Toutefois, c'est bien un élargissement de périmètre qui est proposé dans cet article ; ce n'est pas une suppression des bilans de médication de la convention. L'assurance maladie utilise toujours les termes de « bilans partagés de médication » pour les patients âgés polymédiqués et en tant qu'accompagnement des patients particuliers.

L'accès aux soins leur est donc difficile. Qu'il s'agisse de la dispensation à domicile des médicaments ou du déploiement d'une stratégie de dépistage ou de prévention, il est fondamental que tous les Français puissent y accéder de manière équitable. Cet amendement vise à autoriser les pharmaciens d'officine à se déplacer au domicile des patients, en cas de besoin et dans le respect de leurs missions conventionnelles.

Le Gouvernement a ajouté à l'article 22 un alinéa prévoyant que certaines mesures dépensières de la prochaine convention médicale seront, par dérogation aux dispositions du code de la sécurité sociale, d'application immédiate. Le présent amendement vise à supprimer cet alinéa. Le Parlement sera en mesure de se prononcer sur l'application immédiate de telles mesures

la mise en place d'incitations à l'installation en zones à faible densité médicale. Je mets aux

Les médecins qui s'installent en zone hyperdense- ce n'est peut-être pas la constatation de l'ARS, mais c'est celle de la sécurité sociale -ne peuvent être conventionnés par la sécurité sociale que

l'expérimentation de consultations avancées obligatoires, par des médecins généralistes ou spécialistes, dans les zones sous-dotées. La commission proposera l'adoption de cet article, sous réserve d'une modification tendant à confier l'organisation de ces consultations aux ARS. En cohérence, et pour laisser cette expérimentation être conduite, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dans l'hypothèse

à Montluçon, dans l'Allier, un centre de soins a fermé, laissant 7 000 personnes sans médecin traitant. Malgré une offre de soins parfois pluridisciplinaire et pouvant offrir une couverture complète, les gestionnaires de centres de santé n'ont pas toujours reçu et ne reçoivent toujours pas un appui suffisant. amendement tend donc à renforcer les centres de santé, en permettant la négociation de dispositifs d'aide spécifique dans le cadre de l'accord national des centres de santé.

de cet amendement dans le contexte actuel d'inflation, nous pensons toutefois que celui-ci est déjà largement satisfait. En effet, les accords peuvent prévoir les mesures visant à favoriser l'accès aux soins des assurés, à garantir la qualité et la coordination des soins : modes de rémunération des centres de santé, dispositifs d'aide à l'installation

soignants travaillent dans les établissements de santé genevois, soit 41 % des professionnels du département. Dans l'Ain, 10 % des soignants travaillent en Suisse. La santé est clairement un des secteurs où le travail frontalier est le plus fréquent, pour des raisons évidentes d'écart de salaire. Comme l'a démontré la récente étude étude UFC-Que Choisir, il y a vraiment une fracture sanitaire dans notre pays. Je le vis douloureusement chez moi, comme beaucoup d'entre vous, mais avec, en plus, une situation bien spécifique liée au caractère frontalier

qui dispose : « Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'intérêt de l'extension du coefficient " coût de la vie " pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse. En lien avec ces travaux, une mission a été confiée au préfet de Haute-Savoie pour déterminer des pistes d'évolution en matière de ressources humaines, notamment indemnitaires, qui permettraient de rendre plus attractifs ces territoires. Ces pistes seront potentiellement exportables vers des territoires en difficulté qui ne sont pas transfrontaliers.

partagerez cet avis, monsieur le ministre -que cette évolution dans la répartition des compétences soit préparée, en concertation avec les professionnels concernés et après évaluation des bonnes pratiques et protocoles à retenir.

avec une rémunération- faut-il le rappeler ? -au rabais, et vous comptez sur leur bonne volonté pour exercer dans les zones sous-denses. Cette proposition, que vous avez formulée tout seul, sans concertation avec les syndicats étudiants, ne répondra pas aux problèmes, puisque la nécessité d'être encadré par un médecin senior soulève de très nombreuses questions. Dans les déserts médicaux, quelles seront les perspectives pour trouver un encadrant ? Quelles seront les conditions de travail des internes ? Vous n'y répondez aucunement.

ou d'une mesure de lutte contre les déserts médicaux qui ne dirait pas son nom ? C'est précisément le point de blocage avec les étudiants et les jeunes médecins, alors que cette année professionnalisante faisait plutôt consensus, y compris chez les jeunes

23. Rassurez-vous, il s'agit d'une réforme pédagogique qui est souhaitable- elle était d'ailleurs souhaitée par les étudiants en médecine voilà encore peu de temps -et qui améliorera la réponse aux besoins de santé de demain. C'est d'autant plus important que

C'est également- et cela apparaît peu dans les discussions -la garantie que les étudiants seront thésés avant de commencer la quatrième année. En effet, pour accéder à cette quatrième année de docteur junior, quelle que soit la spécialité, il faut disposer de sa thèse de médecine. Or nous constatons que les étudiants à l'issue de leur formation, la plupart du temps au bout de trois ans, ne sont pas thésés- ils peuvent attendre jusqu'à trois ans pour l'être -, ce qui retarde d'autant plus leur installation. Nous faciliterons l'obtention de la thèse et rendrons ainsi leur installation

l'amendement n° 899. L'article 23 tend à créer une dixième année au cursus universitaire de spécialité médecine générale. Sans concertation avec les organisations syndicales et représentatives, l'introduction dans le PLFSS d'une telle disposition a tout d'une décision unilatérale du Gouvernement. Monsieur le ministre, diriez-vous que les étudiants sont versatiles ? Vous avez dit qu'ils étaient d'accord hier ; pourtant, aujourd'hui, ils sont tous vent debout. Cette disposition, prise dans un contexte national de déficit de médecins généralistes,

Or la formation n'a pas vocation à répondre de manière non structurelle et, qui plus est, non pérenne à des enjeux de maillage territorial et de lutte contre les zones sous-dotées en praticiens. Il s'agit là d'un dévoiement de la formation des futurs médecins.

zones sous-denses. Le résultat probable en termes de des médecins généralistes rend impossibles les parcours de soins coordonnés par un médecin référent, garant de la qualité de l'offre.

C'est une politique malthusienne qui a très bien réussi ! Je crois même qu'en matière d'enseignement supérieur, c'est la politique qui a le mieux réussi. Résultat : il faudrait aujourd'hui inverser complètement la stratégie en redonnant aux

pour les internes en médecine générale, parce qu'ils ne sont pas opposés à avoir une année de professionnalisation ; gagnant par la reconnaissance de leur titre de docteur junior ; gagnant gagnant par un engagement plus fort des médecins généralistes installés pour qu'ils soient encore plus nombreux à être maîtres de stage ; gagnant enfin pour les patients, parce que cela dégagera du temps médical supplémentaire. Il n'y aura pas d'année « blanche » ; je partage l'avis du ministre sur ce point. Le

pratique ambulatoire et pratique à l'hôpital. La question a été évoquée lors de l'examen de la proposition de loi de Bruno Retailleau, mais nous avons fait le choix de réserver le dispositif à la pratique ambulatoire. J'émets donc, à titre personnel, un avis défavorable.

Or le dispositif de la proposition de loi adoptée par le Sénat retient la notion de stage réalisé en autonomie supervisée figurant dans la partie réglementaire du code. Cela implique que le stagiaire consulte seul, mais qu'il doit pouvoir joindre son maître de stage universitaire

associées aux autres modalités d'accompagnement général sont préparées et évaluées par la mission confiée aux quatre personnalités que j'évoquais tout à l'heure, mission qui doit rendre ses travaux à la fin du premier trimestre 2023. De ce fait, je suis défavorable à l'amendement n° 57. Madame Guillotin, je

de voter la proposition de loi de M. Retailleau. Mais ce que vous votez, c'est le projet du Gouvernement, qui permet de demander une quatrième année aux internes de médecine générale pour satisfaire les besoins de l'hôpital. Bien sûr ! Ce que vous êtes en train de créer, c'est une nouvelle catégorie de supplétifs

de la proposition de loi de M. Retailleau. Il est bien évident que l'on ne peut faire de la formation sur une quatrième année de professionnalisation que s'il y a un maître de stage

et laisse le champ libre à la responsabilité de M. le ministre, par le biais de la commission mise en place, pour trouver, dans la concertation, les solutions nécessaires pour rendre cette quatrième année

Vous n'avez avancé aucun argument pour nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la quatrième année de professionnalisation que nous voulons

Peut-être y aura-t-il un exercice mixte en ambulatoire avec le médecin superviseur et des vacations en hôpital. Peu importe ! Ce qu'il faut, c'est que les étudiants en quatrième année soient sur le terrain,

souhaitent les jeunes professionnels. En revanche, vous avez évoqué à plusieurs reprises une « absence de concertation ». Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de concertation ! J'ai commencé à rencontrer les syndicats des étudiants, principalement ceux qui représentent la médecine générale, au mois de décembre 2021,

sur le rapport de notre collègue Bruno Rojouan qui en est issu. Avec cet amendement, nous proposons d'étudier les modalités de mise en oeuvre d'une offre de prévention et de soins itinérante dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante. Pour pallier l'isolement de certains territoires et les difficultés d'accès aux soins amplifiées par la géographie, de nombreuses expérimentations et initiatives ont émergé ces dernières années. Elles se sont particulièrement multipliées avec la crise de la covid-19. Des dispositifs de santé mobile de ce type permettent de se rapprocher des publics les plus fragiles et précaires dans les territoires les plus isolés, où l'accès à la santé est difficile du fait du manque de professionnels de santé.

Guillotin. Les deux premiers alinéas de l'article 24 prévoient la création du guichet unique départemental pour accompagner les professionnels de santé lors de leur installation.

besoin, peut aider à remettre des médecins sur le territoire. La simplification offerte aux jeunes à travers ce guichet unique pourrait convaincre certains et, surtout, accélérer l'installation sur des territoires que, souvent, ils ne connaissent pas.

Elle permet d'avoir un interlocuteur unique, qui offre une approche globale et personnalisée du projet en vue de permettre une agrégation des dispositifs existants.

l'amendement n° 277 rectifié. L'article 24 crée un guichet unique départemental d'accompagnement à l'installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. Le département apparaît comme le meilleur niveau pour organiser l'accès aux soins, la région étant trop éloignée du terrain pour cela. Il est ainsi recommandé de mettre en oeuvre dans chaque département une instance de concertation départementale rassemblant les élus, la CPAM, l'ARS, les professionnels, le conseil de l'ordre, les établissements ainsi que les représentants des médecins et des universités, pour construire des solutions adaptées en fonction du diagnostic territorial et pour aider les professionnels à maintenir l'offre de soins. Cet amendement

dans l'installation de médecins sur leur territoire. Mais, là aussi, il faudrait sans doute s'entendre au préalable sur le rôle du guichet unique et du comité d'aide à l'installation promis par l'étude d'impact. Je ne suis pas convaincue qu'il faille élargir la composition du guichet unique, qui est censé être un

plus âgés souhaitant changer de région ou de département. Par conséquent, je suis défavorable à ces trois amendements.

l'amendement n° 241 rectifié. Les dépassements d'honoraires pratiqués par les médecins conventionnés en secteur 2 constituent un véritable frein à l'accès aux soins pour de nombreux Français, notamment pour les plus modestes. modestes. En zone surdotée ou sous-dotée, des millions de Français n'ont d'autre choix que de consulter des professionnels de santé dont les tarifs dépassent ceux que la sécurité Afin de limiter le recours au dépassement d'honoraires, et ainsi de permettre un meilleur accès aux soins pour les patients, cet amendement tend à priver du bénéfice des aides financières les médecins en situation de dépassement d'honoraires, quel que soit leur lieu d'exercice. L'argent public ne

des dépassements d'honoraires. Or ces pratiques, de la part de médecins conventionnés en secteur 2, constituent un véritable frein à l'accès aux soins pour de nombreux Français, notamment pour les plus modestes. Dans certains départements, les médecins en secteur 1 deviennent de plus en plus rares.

l'Optam, notamment les aides à l'installation. Cela s'inscrit pleinement dans notre objectif d'accès tant financier que territorial à la santé. Il semble néanmoins excessif de prévoir une restriction générale s'appliquant à toutes les aides. Il est important que, selon les dispositifs et l'objectif, le champ de leurs bénéficiaires puisse être adapté au territoire. Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements

préciser que la différence de statut entre exercice en libéral et en centre de santé ne saurait justifier de différence dans l'attribution des aides à l'installation. L'opportunité d'une telle mesure se discute, car il semble

amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Les centres de santé disposent déjà d'aides adaptées à leurs spécificités. C'est le cas notamment de la subvention dite Teulade, qui permet la prise en charge d'une partie des cotisations dues par les centres de santé pour leur personnel. De même, les aides à l'installation destinées aux médecins libéraux ont été transposées pour les centres de santé par l'avenant n° 1 de 2017. Ainsi, un centre de santé installé en zone sous-dense qui emploie trois médecins reçoit une aide de l'assurance maladie de 80 000 euros, soit plus qu'un professionnel libéral. Il est toutefois logique que la somme versée soit dégressive selon le nombre de médecins salariés. Dès lors, si les textes devaient être alignés, les centres de santé perdraient le bénéfice des dispositifs qui leur sont spécifiques, comme la subvention Teulade, et cet amendement ne leur serait pas favorable. Pour ces raisons, le Gouvernement y est défavorable. Je mets